Nous avons mis en lumière que plus de 1,3 million de propriétaires qui habitent leur logement vivent sous le seuil de pauvreté. La propriété ne protège pas de la pauvreté ni de la précarité qui en découle. Nous devons mobiliser des fonds publics pour ne pas laisser les copropriétaires face au fléau du mal logement, y compris en procédant à des acquisitions s’appuyant sur des prêts. La Banque des territoires a chiffré les besoins annuels à environ 9 milliards d’euros. Notre amendement est en deçà de ce montant, puisqu’il vise

qui participent par leurs activités à aggraver le dérèglement climatique – mais ce n’est pas l’objet de cette mission. En revanche, nous avons l’opportunité d’agir pour réduire les émissions de CO2 tout en soutenant le pouvoir d’achat des ménages et des familles, de plus en plus en difficulté pour finir le mois. C’est notamment le cas grâce au dispositif MaPrimeRenov’, qui, en permettant de mieux isoler les logements et de réduire la déperdition énergétique, participe à diminuer la consommation d’énergie et la facture. facture. Malgré l’intérêt de ce soutien à la transition écologique et au pouvoir d’achat, le Gouvernement a souhaité réduire l’enveloppe allouée à MaPrimeRénov’. Nous le savons, il existe 5,8 millions de passoires thermiques où vivent plus de 12 millions de personnes. ces mêmes personnes pourraient mieux vivre si elles ne dépensaient pas une grande partie de leur budget dans les factures d’électricité ou de gaz. Pour respecter nos objectifs, nous devrions rénover 500 000 logements par an, mais nous en atteignons péniblement 65 000. Les 64 millions de tonnes de CO2 émises chaque année par les bâtiments continuent de réchauffer l’atmosphère.

le dispositif MaPrimeRénov’ ne cesse de faire l’objet de coups de rabot d’année en année. Le montant initialement prévu de 4 milliards d’euros a été amputé de 1 milliard d’euros

2,522 millions. Nous apprenons également que Bercy étudierait la possibilité de scinder le dispositif en deux pour une coupe supplémentaire de 700 millions d’euros d’économie. Cette diminution du budget n’est pas acceptable tant elle rend impossible l’atteinte des objectifs nationaux de 370 000 rénovations performantes par an d’ici à 2030 et de 700 000 Alors que la France compte encore des millions de passoires énergétiques, l’effort budgétaire dédié à la rénovation énergétique doit s’inscrire dans le temps, avec des engagements concrets sur la pérennisation des moyens nous permettant d’atteindre nos objectifs, mais aussi de sécuriser l’ensemble d’une filière perpétuellement bouleversée par cette instabilité budgétaire. C’est pourquoi cet amendement vise à maintenir tout simplement le budget alloué à MaPrimeRénov’ à hauteur de 3 milliards afin de conserver un cap clair pour garantir l’efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique. L’amendement

L’assouplissement des critères d’éligibilité à MaPrimeRénov’ courant 2024 et l’apparition d’une dynamique pour les rénovations d’ampleur se sont traduits par une forte hausse du nombre de dossiers déposés.

devraient malheureusement s’intensifier et toucher des territoires jusqu’à présent peu concernés, comme le nord et l’est de la France. Ainsi, 21 millions de logements pourraient être exposés à plus de vingt jours de vague de chaleur dès 2030, contre 9,4 millions actuellement.

Cette inadaptation a des répercussions sanitaires graves, notamment pour les personnes vulnérables – personnes âgées, enfants, etc. Entre 2014 et 2020, la chaleur excessive a entraîné une surmortalité de 33 000 décès d’après Santé publique France. Il est donc urgent d’adapter ces logements,

La prime de transition énergétique MaPrimeRénov’, destinée aux propriétaires pour leur permettre de financer des travaux d’isolation, de chauffage ou encore de ventilation dans leur logement, voit son budget diminuer drastiquement en 2025, après une hausse significative de 2024. Selon nous, cette baisse de crédits au détriment de la transition énergétique affaiblit notre capacité à répondre à des enjeux écologiques, sociaux et sanitaires : réduction de consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, lutte contre la précarité énergétique des ménages et son impact direct sur leur santé.

Les auditions réalisées dans le cadre de la commission d’enquête sur l’efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique, dont j’ai été le rapporteur, ont mis en lumière l’absence de constance, entraînant attentisme et confusion chez les ménages. Au sein du dispositif MaPrimeRénov’, le détail et les conditions des aides changent tous les ans, voire de manière encore plus fréquente. Le service d’accompagnement des particuliers à la rénovation a également changé à plusieurs reprises de mode de financement au cours des dernières années. Afin d’assurer l’efficacité des aides à la transition énergétique, il paraît essentiel d’en garantir la stabilité, en inscrivant la hauteur de leur budget sur le long terme. C’est l’objet de cet amendement d’appel, qui vise à insérer cette stratégie et le volume financier des aides dans une programmation budgétaire pluriannuelle,

que l’on ne peut pas se satisfaire d’un débat qui porte uniquement sur le niveau de l’accompagnement financier de l’État. L’État a fait des choix assez divers ces dernières années.

englobant aussi les C2E, qui servent de manière individuelle aux ménages qui n’ont pas accès à MaPrimeRénov’. Le système reste fragmenté et l’on ne mobilise pas assez les classes moyennes qui ont les moyens de la rénovation.

la sénatrice, la décarbonation du chauffage des bâtiments est essentielle pour atteindre les objectifs climatiques. Néanmoins, des tensions sur la ressource biomasse sont prévues dès 2030, malgré le déploiement d’efforts et de moyens accrus en faveur de la préservation des ressources forestières, de l’isolation et de l’efficacité énergétique. Le Gouvernement a priorisé la stabilité des parcours MaPrimeRénov’ en 2025, afin de faciliter la compréhension et l’adoption par les ménages et les professionnels. Ainsi, les mesures de simplification instaurées au mois de mai 2024 ont été maintenues en 2025 pour soutenir les rénovations des maisons classées F et G dans les diagnostics de performance énergétique. La baisse des barèmes de MaPrimeRénov’ pour les équipements biomasse, de 30 % en moyenne, s’inscrit dans un contexte de nécessaire maîtrise de la dépense publique, tout en permettant de maintenir l’accès aux équipements. Enfin, le bois de chauffage bénéficie d’un taux de TVA réduit à 5,5 %. Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de cet

M. Rémi Cardon. La précarité énergétique s’aggrave dans notre pays. Il est d’ailleurs assez frappant que 37 % des passoires thermiques soient occupées par des ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté.

En témoigne la mission relative à la banque de la rénovation énergétique, lancée à la fin de l’année 2024, à laquelle participent Mmes Margaté et Gacquerre et qui devra proposer des mesures afin d’améliorer le financement du reste à charge des travaux de rénovation, notamment des copropriétés dégradées.

à égalité avec les collectivités locales sur la période 2018 2023. Près de 8 500 logements ont été financés au titre de leur réhabilitation, pour un montant total de subventions d’environ 100 millions d’euros à la fin

mérite légitimement d’être poursuivi. Un engagement de l’État renouvelé en 2025 pour la rénovation des cités minières permettrait, en outre, de se rapprocher, au cours des prochaines années, de la cible initiale de 12 000 logements financés par l’État, par l’État, la rénovation de plus de 2 000 logements supplémentaires. En conséquence, cet amendement a pour objet d’abonder de 8 millions d’euros supplémentaires le programme 135, qui permettra de maintenir le soutien de l’État auprès des collectivités et des bailleurs. Dans le cadre du programme 112 locale » porte la contractualisation de tous les engagements de l’État à l’échelon local. Ces crédits déconcentrés permettent de financer les contrats de plan État région, les contrats de plan interrégionaux État région, ainsi que les pactes territoriaux destinés à financer les priorités locales.

par l’inscription de 100 millions d’euros en autorisations d’engagement et de 25 millions d’euros en crédits de paiement. Madame la ministre, aux questions que les parlementaires du Rassemblement national du Pas de Calais vous ont posées au sujet de l’ERBM, vous avez apporté des réponses différentes selon les cas, me répondant par ailleurs par le mépris, alors même que je ne vous mettais pas en cause. Aujourd’hui, nous sommes à l’heure des actes. Nous demandons, par cet amendement, la concrétisation budgétaire des promesses du candidat Macron dans la réhabilitation des espaces publics des logements du bassin minier. Je le sais, cet effort financier est important, à l’heure où nous recherchons des économies partout pour combler un déficit qui s’est encore creusé de 1 000 milliards d’euros

pour rénover 23 000 logements miniers à vocation sociale très énergivores du Nord et du Pas de Calais, à rénover les espaces publics des cités et à mobiliser un dispositif d’insertion professionnelle des publics résidents. Nous vous rejoignons, puisque, pour concrétiser cet engagement, cet amendement vise à abonder de 8 millions d’euros en autorisations d’engagement et de 2 millions d’euros en crédits de paiement les moyens destinés à cette rénovation.

Malheureusement, les difficultés rencontrées par les Mahorais étaient là avant d’être aggravées par le cyclone Chido, et je crains qu’elles ne perdurent encore tant qu’une intervention publique massive n’aura pas eu lieu. La question de la qualité des logements et de l’accès à ces derniers ne concerne pas que les bidonvilles bidonvilles ou que des personnes en situation irrégulière. D’ailleurs, elle ne concerne pas uniquement Mayotte. À La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, en Nouvelle Calédonie Kanaky, les difficultés de logement sont une réalité, qui s’ajoute à la vie chère et qui contribue à renforcer un sentiment d’abandon. sociaux (Armos) à La Réunion, les logements de plus de 20 ans nécessitant une remise à niveau représentent la moitié du parc locatif social, soit plus de 35 000 logements.

à la réhabilitation du parc privé en outre mer en accompagnant les ménages ultramarins par des aides financières. Entre 2017 et 2022, plus de 25 000 logements ont ainsi été traités.

le Gouvernement ne peut prétendre atteindre les objectifs de rénovation qu’il a fixés sans en donner les moyens aux bailleurs sociaux. C’est pourquoi, conformément aux travaux de la commission d’enquête sénatoriale sur l’efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique, nous avons proposé d’allouer, dès 2024, 1,5 milliard

sa participation au 83 congrès HLM en annonçant notamment la création d’un fonds de 1,2 milliard d’euros pour la rénovation du parc social, soit 400 millions d’euros

contrairement à l’Hexagone. Cela crée une rupture d’égalité que nous ne pouvons plus ignorer. Ce sont précisément 217 000 familles ultramarines qui sont concernées. Le différentiel du forfait charges est

reprises à Paris, ou celles de 2009 en Guadeloupe, les populations ultramarines pâtissent de la cherté de la vie. Les écarts de prix entre l’outre mer et l’Hexagone atteignent jusqu’à 40 % pour les produits alimentaires et près de 20 % pour l’énergie. Ces disparités, déjà relevées par l’Insee il y a plusieurs années, se sont amplifiées avec l’inflation. En parallèle, les revenus de ces territoires sont structurellement plus faibles, aggravant les situations de précarité et les inégalités sociales. Le taux de pauvreté est significativement plus élevé que dans l’Hexagone, tout comme celui du chômage, qui affecte particulièrement les jeunes générations. Le barème des aides au logement, bien que calqué sur celui de l’Hexagone, reste actuellement

pour supprimer le mois de carence pour l’ouverture de ce droit. La contemporanéisation des ressources représente à la fois une modernisation et une économie importante. Il serait donc parfaitement justifié, dans le cadre d’une simplification et d’une mise à jour du dispositif, et afin de renforcer son équité, de supprimer une mesure qui est une source d’incompréhension et de colère pour les ménages modestes s’installant dans un nouveau logement.

Mme Viviane Artigalas. Cet amendement vise à rétablir l’APL accession pour un montant estimé à 50 millions d’euros. L’APL accession constitue un outil très efficace pour aider les ménages modestes à accéder à la propriété dans un contexte où les conditions d’octroi des prêts

avec une grande efficacité, notamment le PTZ, les taux réduits de TVA pour des travaux de construction ou d’achat sous conditions de ressources, le prêt social location accession (PSLA)

la loi de finances pour 2018 a prévu l’extinction pour les prêts signés à compter du 1 janvier 2018. Ce dispositif était en forte décroissance,

Parmi les personnes qui rencontrent des difficultés pour accéder au logement figurent celles qui, malgré leur travail, ne peuvent se loger. Un quart des personnes sans domicile fixe occupent un emploi. Cet amendement s’appuie sur les travaux de la Fondation Abbé Pierre, ainsi que sur les retours de bailleurs et de maires, qui constatent la difficulté de loger des demandeurs, dont le taux d’effort est de plus en plus important. Ce taux, calculé pour vérifier que le loyer ne dépasse pas un tiers des ressources du demandeur, afin d’assurer sa solvabilité,

du Gouvernement ? Cet amendement vise à créer un fonds national d’aide à la quittance, doté de 200 millions d’euros, pour faciliter l’accès au parc social des ménages disposant de faibles revenus. Le droit au logement opposable (Dalo) garantit l’accès de tous à un logement social, y compris aux personnes les plus modestes.

Le scrutin est ouvert.

Depuis 2021, les Ccapex et les équipes mobiles jouent un rôle central dans la lutte contre les expulsions locatives et dans la recherche de solutions de relogement pour les ménages en difficulté.

les Ccapex en sont réduites à traiter un nombre marginal de dossiers, très faible au regard du nombre d’assignations dans les territoires concernés. Même dans les départements les plus performants, les ratios entre situations étudiées et assignations en justice restent inférieurs à 20 %. Au total, sur l’échantillon analysé par la Cour des comptes, le nombre de dossiers étudiés par les Ccapex n’a que faiblement augmenté, passant de 2 250 en 2016 à 2 736 en 2021. Il s’agit donc d’un enjeu extrêmement important. Si l’on ne veut pas engorger les tribunaux, donner plus de moyens aux Ccapex permettrait de résoudre

de novembre dernier, la loi de fin de gestion a ajouté 250 millions d’euros au programme afin de prendre en charge les 203 000 places d’hébergement confirmées par Mme la ministre, le

Le ministère des finances sous dote ce programme à hauteur de 280 millions d’euros, alors même que la Cour des comptes recommande à l’État de garantir aux gestionnaires des centres d’hébergement une trajectoire

le programme 177 a fait l’objet d’un effort budgétaire important ces dernières années pour répondre à la croissance des besoins.

de poursuivre le travail pour améliorer la qualité du service rendu aux personnes hébergées, tout en renforçant la performance sociale du dispositif. Le plan Logement d’abord reste en particulier une priorité pour accélérer l’accès au logement, diminuer la durée des séjours en hébergement, voire permettre l’accès direct au logement depuis la rue. En conséquence, le Gouvernement abondera autant que nécessaire ce programme en cours d’année, de manière à faire face aux éventuelles impasses de financement

environ 3 000 femmes et presque autant d’enfants sans abri passent la nuit dans la rue. Le rapport d’information indique que, pour gérer la pénurie de places, certaines préfectures ont défini des critères de plus en plus stricts

d’agressions sexuelles. Les acteurs associatifs sont unanimes : il n’est pas une femme sans abri rencontrée ou accueillie par leur structure qui n’ait été victime de violences dans la rue.

que, conscient des vulnérabilités accrues auxquelles les femmes sans domicile sont confrontées, l’État a mis en place des dispositifs spécifiques pour améliorer la prise en compte de leurs besoins dans le cadre du pacte des solidarités 2023 2027. Quelque 1 500 places d’hébergement destinées aux femmes enceintes ou en post maternité ont été pérennisées, portant le parc national à un total de 2 500 places.

qui a été tuée, poignardée dans sa voiture, parce qu’elle tentait de trouver des solutions face à un conjoint violent. Dans le cas de Chloé, la plainte et la fuite

Ces amendements attestent la sensibilité transpartisane qui anime cet hémicycle au regard de la détresse que connaissent ces femmes et ces enfants dans la rue, dans leurs maisons, partout dans notre société.

je vous remercie,

Au regard des conclusions de ce rapport d’information, il paraît impératif de proposer des solutions d’hébergement en aval des maternités pour accueillir les populations les plus précaires. Cet investissement social doit être pensé en coordination entre l’État, compétent en matière d’hébergement d’urgence, et les départements, compétents pour l’hébergement des femmes enceintes et des mères isolées avec des enfants de moins de 3 ans.

Fort des résultats obtenus, le Gouvernement a décidé de pérenniser le dispositif, en 2024, pour l’ensemble du quinquennat, le Pacte des solidarités. Cette mesure est complétée par le financement de 50 places de Lits halte soins santé pédiatriques pour des mères dont les nourrissions nécessitent un accompagnement médical renforcé dans la durée.

Le Gouvernement a confirmé son soutien aux SIAO et aux acteurs de la veille sociale en 2024, en leur allouant un renfort de 500 équivalents temps plein, soit 25 millions de crédits supplémentaires, dans le cadre du second plan Logement d’abord. Au total, les effectifs atteignent aujourd’hui 2 100 ETP, soit quasiment un doublement par rapport à l’effectif de 2017. L’année 2025 doit permettre de tirer les bénéfices de ces recrutements nouveaux en matière d’« aller vers », d’amélioration des évaluations sociales, d’accélération et d’adaptation des orientations des publics accueillis. Ainsi, il paraît prématuré d’engager de nouvelles mesures de renfort, mais nous suivrons,

afin de rétablir le niveau de financement de l’année précédente. Le plan quinquennal Logement d’abord a montré son efficacité en permettant à des personnes en situation de précarité d’accéder à un logement pérenne, réduisant ainsi la dépendance à l’hébergement d’urgence. L’intermédiation locative représente donc un levier crucial pour renforcer l’offre sociale dans le parc privé en garantissant un accompagnement adapté aux ménages exclus de l’offre classique.

tout à fait insatisfaisant, pour ne pas dire plus. L’accompagnement social des ménages est, nous le savons, un facteur clé permettant de garantir l’accès et le maintien dans le logement. Depuis le pic atteint en 2021, l’État s’efforce, en lien avec l’ensemble des parties prenantes, de réduire le nombre de places à l’hôtel au profit de solutions plus qualitatives. La question de l’accompagnement est cruciale dans cette orientation. En conséquence, le parc de places à l’hôtel a diminué de 15 % pour atteindre 64 300 places, fin de 2024. En 2024, l’État a investi à hauteur de 378 millions d’euros dans l’accompagnement social des publics dans l’hébergement généraliste, étant consacrés à l’accompagnement des ménages à l’hôtel. L’accès au logement social a également été un axe d’action très important. Ainsi, depuis 2018, plus de 122 000 attributions

Mme Annie Le Houerou. Cet amendement vise à compenser les financements non perçus par les établissements associatifs d’accueil, d’hébergement et d’insertion au titre des revalorisations salariales Ségur annoncées en 2024 et non versées à date. La mobilisation du secteur médico social a permis l’obtention d’un agrément

du Gouvernement ? Le secteur du travail social traverse une crise importante d’attractivité et l’État s’est à plusieurs reprises fortement engagé,

et du logement. Quelque 144 millions d’euros sont désormais consacrés annuellement au financement de cette mesure pérenne. Ensuite, la hausse du point d’indice dans les conventions collectives de la branche de l’action sanitaire sociale et médico sociale à but non lucratif

soient payées aux salariés concernés dès l’année 2024, ce qui devrait apaiser vos inquiétudes. Le solde des crédits dus aux employés au titre de 2024 sera versé en 2025 dès le déblocage des reports de crédits. Cette mesure continuera d’être financée en 2025 dans le cadre du budget

était de 2,2 % en moyenne en 2024, pèse lourdement sur la charge des associations gestionnaires et crée des situations de déficit structurel qui ne sont pas tenables à moyen terme.

Dans le même temps, les acteurs de terrain constatent une augmentation de la précarité et des besoins d’accompagnement des personnes qui se retrouvent dans une telle situation. Afin de répondre à ces deux enjeux,

sociale (CHRS) depuis 2023. La lutte contre la précarité alimentaire passe aussi par la rénovation et l’adaptation des structures d’hébergement. Depuis 2008, l’État finance, le programme d’humanisation et de réhabilitation des structures, qui intègrent la possibilité de cuisiner. Entre 2017 et 2022, ce programme a permis la rénovation de près de 4 500 places et 141 structures, pour un budget global de plus de 50 millions d’euros. Enfin, l’État porte une attention particulière à la situation des personnes hébergées à l’hôtel, où l’on note une prévalence élevée d’insécurité alimentaire liée à l’absence de prestations repas et au manque d’équipements. En 2021, l’État a soutenu la création de plus de soixante tiers lieux alimentaires, à hauteur de 25 millions d’euros sur deux ans. Ces lieux permettent aux familles hébergées à l’hôtel d’accéder à des équipements de cuisine pour préparer leur propre repas. En juillet 2022, plus de 12 000 personnes ont pu bénéficier de ces structures. Fort de ces résultats, le Gouvernement a décidé de pérenniser ces tiers lieux dès 2024

Près de 20 % des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté ; 46 % d’entre eux travaillent pendant l’année scolaire ; et plus de la moitié estiment que leur travail est indispensable pour s’en Le logement représente leur premier poste de dépenses : 60 % en moyenne de leur budget en 2022. Or la production de logements étudiants est en baisse depuis 2017

Surtout, le Premier ministre a annoncé la construction de 15 000 logements par an, pendant trois ans, grâce à la mobilisation du foncier disponible de l’État. Je crois beaucoup à la mise à disposition du foncier public,

Cette aide est absolument nécessaire. Il est vital d’encourager les maires à autoriser les permis de construire et à accompagner les opérations de production de logements, en les aidant à financer les équipements nécessaires à l’accueil de nouveaux habitants. Conformément à l’annonce faite cette semaine par le Premier ministre, le Gouvernement déposera un amendement

des difficultés financières en plein cœur de la phase opérationnelle du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), dont le prolongement ne serait par conséquent plus soutenable à moyen terme. Je rappelle que les crédits budgétaires prévus par la loi de finances initiale

Ce manquement de l’État à ses engagements risque de placer l’Anru dans une situation de déficit en 2027, rendant difficile l’exécution des objectifs qui lui ont été assignés, alors même que le nouveau programme de rénovation urbaine est un succès.

une montée en puissance opérationnelle et financière. À la fin de 2024, 2,1 milliards d’euros de subventions avaient été engagés au titre de 2024 et 975 millions d’euros avaient été mis en paiement. Cela porte le montant des engagements cumulés à plus de 9,2 milliards d’euros de subventions et celui des paiements cumulés à plus de 2,75 milliards d’euros.

Il est donc urgent,, de rétablir ces financements et de donner aux acteurs des quartiers populaires les moyens de mener une politique solidaire de lutte contre les inégalités. Ainsi, nous proposons d’augmenter de 90 millions d’euros les moyens de la politique de la ville.

Les économies ne doivent pas se faire sur le dos des plus pauvres, alors qu’ils subissent déjà de plein fouet une inflation galopante et que l’action publique est plus que jamais nécessaire pour ne pas aggraver la cassure qui s’opère dans certains territoires de la République. Quel est l’avis de la commission ? La commission émet

que les crédits votés l’an dernier étaient déjà insuffisants pour financer en année pleine les 6 514 postes ouverts. La baisse des crédits en 2025 augure donc d’une nouvelle baisse des effectifs, quand bien même il est souhaitable de développer les actions de médiation dans l’éducation, les transports, la santé et la tranquillité publique. Il est également nécessaire de conforter la logique d’insertion sociale et professionnelle au bénéfice des titulaires de contrats adultes relais. Cet amendement vise donc à abonder le

une série de mesures avaient été annoncées, dont la généralisation des cités éducatives. Pourtant, les crédits alloués aux cités éducatives sont en baisse. L’annonce d’un prochain CIV est certes

ces bataillons ont permis le recrutement d’éducateurs spécialisés et de médiateurs sociaux dans des quartiers ciblés, dits de reconquête républicaine. L’objectif était de prévenir la délinquance juvénile et de renforcer les liens sociaux entre habitants,

dans ce secteur dynamique. Toutefois, le montant de l’aide au poste n’a pas été revalorisé depuis plus de vingt ans. Aujourd’hui fixé à 7 164 euros par an, il ne représente plus 17 % d’un salaire. La situation n’est plus tenable, tout particulièrement dans nos territoires ultramarins,